sur l'action n° 01 du programme 122, « Concours spécifiques et administration ». Cette action ne comprend que 94 millions d'euros en autorisations d'engagement. Or l'adoption cumulée de ces amendements conduirait à prélever sur ses crédits une somme supérieure. En conséquence,

M. Didier Marie. Cet amendement vise à revaloriser de 50 millions d'euros les crédits de la dotation politique de la ville, la DPV, pour atteindre un montant de 200 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 161 millions d'euros en crédits de paiement.

l'amendement n° II-670 rectifié. La DSIL a, depuis sa création en 2016, apporté la preuve de sa pertinence dans la concrétisation des projets d'investissement engagés par les communes et les EPCI. Elle n'est d'ailleurs pas étrangère au redressement des investissements du bloc communal enregistré ces années, après plusieurs années de baisse dues notamment aux diminutions de la DGF. La loi de finances pour 2018 avait déjà procédé, sous couvert de modifications des concours des programmes 119 et 122, à une diminution des crédits de la DSIL. Elle avait aussi permis, reconnaissons-le, de pérenniser cette dotation.

La « maquette LOLF » nous contraint à financer cette augmentation par une diminution correspondante des crédits de l'action n° 01, « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122. Malgré certains écueils- je pense notamment à une sous-consommation des crédits, que je trouve d'ailleurs étrange étrange au vu du nombre de projets engagés par les communes et les intercommunalités -, nous estimons que la DSIL doit être maintenue, comme l'est notamment la DETR, et que le fragile édifice du soutien à l'investissement public local doit être préservé.

des communes éligibles. Cette enveloppe supplémentaire serait financée par les collectivités elles-mêmes. Il nous semble que la fin du plafonnement ne serait pas de nature à déstabiliser la DPV, puisque 19 communes supplémentaires seraient éligibles

a déjà été majorée de 8 millions d'euros en 2018. Dans la mesure où l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques résulte d'une décision facultative des communes, il ne nous semble pas opportun d'aller au-delà, d'autant que du présent amendement se traduirait par une diminution des crédits consacrés aux aides exceptionnelles aux collectivités territoriales, voire par une baisse de la DGF ou des variables d'ajustement. Je demande donc également de retrait

et les crédits d'investissement pour les communes. Cela nous oblige aujourd'hui à arbitrer entre la DPV et la DSIL,

Monsieur Raynal,

CFL. L'amendement tend, d'une part, à prévoir des remplaçants et, d'autre part, en cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un membre élu du Comité, à autoriser l'association nationale d'élus locaux représentative à désigner un nouveau membre jusqu'aux élections suivantes.

des différentes catégories de collectivités territoriales. Compte tenu des obligations importantes incombant aux exécutifs des collectivités, il paraît nécessaire de leur permettre de se faire représenter par un de leurs adjoints ou de leurs vice-présidents, en vue d'assurer un fonctionnement optimal du comité des finances locales. En outre, cet amendement tend également à instaurer une procédure visant à ouvrir la possibilité de pourvoir les sièges laissés vacants en cas de décès

Aujourd'hui, le pacte de stabilité financière s'applique aux communes ne dépassant pas le seuil de 150 000 habitants, ce qui nous semble déraisonnable.

Pour ces dernières, de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à celui des communes de la même strate et dont la part des résidences secondaires est supérieure à 30 %, la population DGF serait majorée de 1,5 habitant par résidence secondaire, au lieu de un actuellement. Le montant estimé de cette mesure est contenu à environ 7 millions d'euros. Toutefois, ce dispositif ne permet pas de répondre aux difficultés rencontrées par certaines communes, notamment certaines petites stations de montagne. Ces dernières, qui comptent un grand nombre de résidences secondaires et qui connaissent donc de fortes variations saisonnières de population, doivent mettre en place des équipements et des infrastructures adaptés occasionnant un surcoût parfois très important. Pour ces communes souvent isolées, le secteur touristique constitue une composante essentielle de l'activité économique. Le bulletin d'information statistique de la DGCL, la direction générale des collectivités locales, de janvier 2017 relevait d'ailleurs que les dépenses de fonctionnement étaient plus élevées dans les communes touristiques ou de montagne comptant un grand nombre de résidences secondaires et que, parmi ces dernières, les dépenses étaient plus élevées encore dans les petites communes, notamment dans les petites stations de sports d'hiver. Ces deux amendements visent à tirer les conséquences de cette situation. Leurs auteurs prévoient de majorer la majoration de population DGF en la portant à deux habitants

concernées étant au demeurant limité, cette modification aurait des conséquences insignifiantes à l'échelle de l'enveloppe DGF. L'adoption de ces assouplissements permettrait à certaines communes de mieux faire face aux importantes et particulières contraintes qui pèsent sur elle.

la population DGF, laquelle correspond à la population INSEE majorée d'un habitant par résidence secondaire et par place de caravane. Cette majoration est portée à deux habitants pour les communes éligibles, l'année précédente, à la DSU ou à la DSR fraction bourg-centre.

rapporteur spécial. Le présent amendement vise à préciser que le potentiel fiscal pris en compte pour déterminer l'éligibilité de certaines petites communes touristiques à la sur-majoration de leur population est celui qui est connu au 1 janvier de l'année précédant la répartition.

La contribution au redressement des finances publiques est supprimée.

voient un certain nombre de charges en fonctionnement et en investissement peser sur leur budget, certes avec des recettes réelles de fonctionnement par habitant supérieures à la moyenne. Je pense aux opérations d'intérêt national.

des décisions passées.

verticale à la place de celles qui ont le plus de moyens. En effet, chaque année, la dotation forfaitaire des communes est écrêtée pour financer des contraintes internes à la répartition de la DGF, en particulier la progression des dotations de péréquation. Afin de ne pas faire supporter la charge de cette minoration par les communes les moins favorisées, qui ont vocation à bénéficier pleinement de la hausse des dotations de péréquation, la loi prévoit que l'écrêtement est réalisé sur la dotation forfaitaire des communes qui présentent un certain niveau de potentiel fiscal par habitant. Ce sont ainsi les communes dont les dotations forfaitaires sont les plus élevées qui financent la progression de la péréquation pour les communes les plus en difficulté. Toutefois, la contribution au redressement des finances publiques a minoré la dotation forfaitaire des communes, voire fait disparaître la dotation de certaines d'entre elles. Ces communes, qui sont donc en situation de DGF négative, échappent au financement de la progression des dotations de péréquation, alors même qu'elles peuvent présenter un niveau de richesse très élevé, qui se traduit par un potentiel fiscal par habitant élevé, lequel peut être quinze fois supérieur au seuil d'écrêtement. Il paraît donc nécessaire de remédier à cette situation en faisant participer ces communes au financement de la péréquation verticale. À l'image de la contribution au redressement des finances publiques, l'écrêtement calculé pour ces communes prendrait la forme d'un prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité. telle évolution permettrait d'assurer une plus grande solidarité entre les collectivités et de mieux répartir la charge entre les communes écrêtées.

La hausse continue de la péréquation verticale permet d'assurer la croissance de la DGF des communes fragiles. Or de nombreuses communes voient leur DGF stagner, voire diminuer, en raison de l'écrêtement appliqué à la dotation forfaitaire. Ces effets contre-péréquateurs de l'écrêtement sont fortement accentués dans les communes des DOM qui bénéficient de l'octroi de mer. Par ailleurs, celles qui subissent une hémorragie démographique et qui, de ce fait, présentent un potentiel financier par habitant artificiellement élevé sont doublement pénalisées. pénalisées. Le montant de l'écrêtement ne peut être supérieur à 1 % des recettes réelles de fonctionnement, recettes de l'octroi de mer comprises. En 2017, la Cour des comptes s'était étonnée que l'on intègre l'octroi de mer dans l'assiette pour limiter l'écrêtement,

vise uniquement à retraiter du panier des recettes réelles de fonctionnement des flux pour lesquels ces trois communes ne servent que de boîte postale. Quel est l'avis de la commission ? Vous savez,

La baisse des dotations aux collectivités résultant des derniers budgets a des répercussions catastrophiques et coûteuses sur le long terme dans les territoires les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle la contribution au redressement des finances publiques a été assortie d'un renforcement significatif de la péréquation nationale ciblé sur les territoires les plus fragiles, afin de compenser la baisse de leurs dotations. Malheureusement, ce principe de solidarité nationale n'a pu être respecté pour les communes des départements et régions d'outre-mer, les DROM, en raison d'un système de péréquation nationale particulièrement désavantageux pour les outre-mer. En effet, ce sont plus de 60 % de la CRFP des communes ultramarines qui n'ont pas été compensés, alors que pour les 10 280 communes cibles de la DSU et de la DSR, la CRFP a été intégralement compensée par la hausse de la péréquation. Comment justifier un tel écart de traitement pour des communes qui, si elles n'étaient pas dans les outre-mer, auraient été éligibles à la DSU et à la DSR ? Il en résulte que les investissements des communes des DROM chutent de manière vertigineuse- moins 25 % contre 0,6 % au plan national en 2016 -, et la hausse de la fiscalité atteint des records- 8 % contre 1,2 % à l'échelon national faisant le lit de nouvelles explosions sociales en cours et à venir. Dès lors que la Cour des comptes a relevé une différence de traitement non justifiée à l'égard de où la dotation de péréquation verticale moyenne par habitant est de 75 euros, contre 125 euros pour les communes de l'Hexagone qui y sont éligibles, soit un manque à gagner de 137 millions d'euros au total pour l'outre-mer- 42 millions d'euros pour les COM, les collectivités d'outre-mer -, la responsabilité nationale, plus que la solidarité nationale, impose des mesures rectificatives d'urgence. Face à ce constat, le Gouvernement prépare pour l'année prochaine une réforme des dotations pour les communes ultramarines. Mais nous devons agir dès maintenant. Le retard accumulé depuis la mise en place de la CRFP ne sera jamais rattrapé. Faisons au moins en sorte qu'il ne continue pas à s'accroître. C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de limiter de moitié le retard des communes d'outre-mer sur les communes de l'Hexagone éligibles à la péréquation verticale, ce qui permettrait de neutraliser globalement la contribution des 112 communes des DOM. Quel est l'avis de la commission ? La

et je reçois toujours la même réponse. La Cour des comptes a constaté qu'il y avait une discrimination, une inégalité, à l'encontre des outre-mer. Mais régulièrement, on nous renvoie vers le CFL, lequel nous renvoie

La montée en puissance de ces deux dotations de péréquation verticale est continue depuis plusieurs années. La DSU s'établit à plus de 2 milliards d'euros en 2018. Les différentes composantes de la DSR la portent à 1,5 milliard d'euros Cette progression a été de 180 millions d'euros en 2017 pour chacune de ces deux dotations. L'an passé, elle n'a été que de 110 millions d'euros pour la DSU, grâce à l'adoption d'un amendement, et de 90 millions d'euros pour la DSR. Le présent projet de loi de finances ne prévoit, à ce stade, qu'une augmentation de 90 millions d'euros pour chaque dotation. On peut donc s'interroger sur les mécanismes d'éligibilité à ces dernières. Nous devrons d'ailleurs examiner les amendements prévoyant des garanties en cas de sortie, je pense notamment à la fraction bourg-centre de la DSR. Une éventuelle refonte de la DGF nécessiterait de se pencher sur ces problématiques. Cependant, on ne saurait, dans l'attribution de la DGF, nier l'importance de la prise en compte de critères sociaux et des contraintes particulières qui pèsent sur les communes rurales ou peu riches. Pour ces raisons, estimant que la trajectoire de progression de la DSU et de la DSR doit être soutenue, nous souhaitons que la revalorisation soit portée à 110 millions d'euros

lieu de 90 millions d'euros. Pour rappel, lors du quinquennat précédent, des efforts substantiels ont été réalisés pour réduire les inégalités entre communes, qu'elles soient éligibles à la politique de la ville ou qu'elles soient rurales. En 2016 comme en 2017, la DSU la DSR ont progressé de 180 millions d'euros. L'an dernier, une discussion a eu lieu : le Gouvernement a proposé 90 millions d'euros et, après débat, a considéré que le montant de 110 millions d'euros était le minimum qu'il fallait assumer,

a été refusée, mais nous restons cohérents avec la ligne que nous avons défendue. Je rappelle que, l'an dernier, le montant supplémentaire de DSU et de DSR

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination de l'éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale. Malgré une population permanente inférieure à 1 500 habitants, les communes visées supportent en effet des charges de centralité importantes. La perte de leur fraction bourg-centre menace aujourd'hui la pérennité des services publics de proximité qu'elles doivent assurer. Par ailleurs, ce plafonnement a entraîné un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne. Lors des débats du projet de loi de finances pour 2018, il avait été convenu que ce sujet serait traité dans le cadre de la future réforme de la DGF. Dans combien d'années ? Cette dernière n'étant pas encore à l'ordre du jour, il paraît d'autant plus urgent de supprimer cette mesure inéquitable pour les communes concernées par le plafonnement introduit par la loi de finances pour 2017. J'ajoute que cela ne créera en rien

l'objet porte sur la fraction bourg-centre de la DSR. Cette fraction reconnaît le rôle de centralité que jouent un certain nombre de bourgs ruraux grâce à l'existence d'équipements et de services. Dessinée à gros traits, la carte des communes concernées correspond au maillage des anciens chefs-lieux de cantons ruraux. La loi de finances pour 2017 a instauré un plafonnement de population pour l'éligibilité à la DSR bourg-centre basé sur la population DGF. Cette disposition a entraîné pour les communes concernées une diminution de l'attribution perçue au titre de la DSR bourg-centre, voire la perte d'éligibilité à cette dotation. Cela concerne principalement les petites communes touristiques comptant un grand nombre de résidences secondaires. L'amendement n° II-675 rectifié vise à supprimer le plafonnement introduit en 2017. Pour rappel, un tel amendement a été adopté par notre sage assemblée l'an est un amendement de repli : il tend à proroger le mécanisme permettant à une commune perdant l'éligibilité de percevoir une garantie de sortie égale à 50 % du montant perçu en 2016. Cette garantie de sortie, créée en 2017, a été prorogée dans la loi de finances pour 2018.

vous savez qu'il a été mis en place et introduit sur l'initiative de notre collègue député Joël Giraud, que l'on ne peut pas soupçonner de manquer de considération pour les communes touristiques. Lors de l'examen de la loi de finances pour 2017, les députés ont prévu de viser la population DGF au lieu de la population INSEE, pour favoriser les communes touristiques,

accorder une nouvelle année de garantie supplémentaire aux communes touristiques lorsqu'elles perdent la DSR, une telle disposition revient à leur accorder une garantie trois fois supérieure à celle des autres communes.

sous couvert de gestes et de preuves d'amour pour la ruralité, on parle de quelques communes- ô combien importantes à votre coeur -qui sont souvent de montagne, petites et touristiques.

Cet amendement vise à limiter le financement de l'enveloppe de 30 millions d'euros supplémentaires pour la dotation d'intercommunalité par les minorations internes au sein de la dotation globale de fonctionnement à la moitié de cette enveloppe, soit 15 millions d'euros, en accord avec les conclusions du comité des finances locales. En effet, les travaux du CFL sur la réforme de la dotation d'intercommunalité ont, à l'unanimité, conclu à la nécessité d'augmenter cette dernière de 30 millions d'euros, afin non seulement de permettre à tous les EPCI à fiscalité propre de toucher une fraction de cette dotation, mais également d'atténuer les effets de la réforme. Sur

? Monsieur le sénateur Marie, par ces amendements, vous demandez en quelque sorte pardon d'avoir diminué la DGF pour l'ensemble des communes et des départements de France ces cinq dernières années. Vous qui avez

de celles et ceux qui contribuent aux équilibres budgétaires, nous ne l'avons pas fait de gaieté de coeur. Je l'ai souligné dans mon propos liminaire

La situation n'est plus la même. C'est la raison pour laquelle nous pensons que nous pouvons prendre un certain nombre de dispositions permettant de rééquilibrer la situation de nos collectivités, tout en insistant sur la péréquation que nous avons mise en oeuvre sous le quinquennat précédent, que nous souhaitons poursuivre aujourd'hui et qui nous paraît utile et indispensable pour bon nombre de nos communes.

En effet,, il n'y a qu'un seul citoyen, le citoyen contribuable, et qu'une seule dette, la dette de la nation française dans son ensemble. Certes, on peut opposer les finances locales aux finances nationales-

pour le savoir. Arrêtons ce petit jeu et faisons enfin autre chose que cette politique qui consiste à déplacer des virgules d'un endroit à un autre en gardant exactement le même système. Je n'ai pas de conseils à donner, mais, si vous faites

Le projet de loi de finances pour 2019 modifie les règles de fixation de la dotation d'intercommunalité pour tous les EPCI à partir du 1 janvier 2019. Le montant de cette dotation ne sera plus lié au statut, mais sera modulé selon le degré d'intégration de l'EPCI.

Certains EPCI ont donc engagé un processus de transformation en un EPCI relevant d'une nouvelle catégorie. Ces décisions de transformation ont notamment entraîné le transfert des compétences nécessaires pour relever de la nouvelle catégorie à partir du 1 janvier 2019. L'ensemble de l'argumentation pour changer de statut a été développé bien avant que ne soient connues les nouvelles règles édictées par ce projet de loi de finances. présent PLF, ces EPCI sont perdants financièrement pour ce qui concerne la dotation d'intercommunalité. Leur dotation est liée non plus au statut, mais à leur niveau d'intégration mesuré par le coefficient d'intérêt fiscal sur la base du niveau de la dotation d'intercommunalité 2018,

plus importante. Nous pensons qu'en 2019, date d'entrée en vigueur de la réforme, tous les EPCI doivent être soumis aux mêmes critères. En même temps, techniquement, la mesure que vous proposez n'est pas si simple, car, pour mon cher collègue, il conviendrait de procéder d'abord à une répartition fictive de la dotation d'intercommunalité 2019 à partir des critères de 2018 et de refaire ensuite mouliner la machine : cela paraît assez complexe. Selon vous, les EPCI qui changent de catégorie sont perdants. Ce n'est pas certain.

était attendue et il s'agit de faire preuve de souplesse, même de bienveillance, à l'égard des structures qui vont évoluer juridiquement. Ce qui a été imaginé

Favorable

étudiée dans le cadre du comité des finances locales ; elle conduirait à de très importantes pertes pour les communautés d'agglomération, alors même que cette catégorie d'EPCI a particulièrement souffert des dysfonctionnements des enveloppes de la dotation d'intercommunalité. La commission demande donc aux auteurs de ces deux

Le coefficient d'intégration fiscale a été créé pour encourager un certain niveau d'intégration administrative et financière entre communes et intercommunalités, et ceci, à l'origine, en 1999- j'en ai quelques souvenirs -, pour éviter les communautés de pure redistribution. Aujourd'hui, cette préoccupation ne pèse plus vraiment. Et je fais observer que si l'on ne plafonne pas le coefficient d'intégration fiscale à un certain niveau, l'objectif, dans une perspective d'optimisation, tout ceci se passant naturellement à somme nulle-

Lorsqu'une communauté de communes a été créée, lorsqu'elle rassemble, donc, des communes appartenant à divers EPCI, ceci sans succéder à l'un de ces EPCI, aucune garantie spécifique de stabilité de la DGF n'est prévue. Une garantie a pourtant été instituée pour les communautés d'agglomération créées, qui, lors de leur deuxième année d'existence, ne peuvent pas voir leur dotation baisser par rapport à celle de l'année précédente. Cette carence dans les mécanismes très complexes de garantie applicables au calcul de la dotation d'intercommunalité a eu un impact significatif sur la dotation dont ont bénéficié deux communautés de communes à fiscalité professionnelle unique en 2018.

par l'évolution de leurs indicateurs individuels - seules la contraction des enveloppes et l'absence de garantie les ont pénalisées, alors que les autres communautés de communes ont toutes bénéficié de mécanismes,

sans pour autant leur redonner un niveau d'attribution comparable à celui de 2017. Il est ainsi proposé de déplafonner la progression dont elles bénéficieront en 2019. Cet avantage se justifie par la situation très particulière de ces deux communautés de

de subsidiarité. À la suite de la refonte de la carte intercommunale, de nombreux EPCI à fiscalité propre, devenus extrêmement vastes, ont été conduits à restituer des compétences de proximité à leurs communes membres,

baisser le coefficient d'intégration fiscale des EPCI concernés et, partant, leur dotation d'intercommunalité. Ce choix de réorganiser les compétences locales, guidé par le principe de subsidiarité, s'est donc traduit par une perte nette de ressources pour les territoires concernés pris dans leur ensemble. Afin de résoudre cette difficulté liée à la structure même de la dotation d'intercommunalité, notre amendement vise à ce que, en cas de baisse du CIF d'un EPCI à fiscalité propre, la somme correspondant à la diminution de dotation qui en résulte vienne financer une dotation de consolidation répartie entre les communes membres au prorata de leur population. Ainsi, les élus locaux pourront ajuster la répartition des compétences au niveau local en fonction des nécessités du terrain, au lieu de se déterminer selon des considérations purement financières.

à l'intérieur d'une grande intercommunalité, on y perde des dotations,

quoi qu'on pense de cette réforme de la dotation d'intercommunalité, elle a été largement négociée par et avec toutes les associations d'élus, et avec le comité des finances locales, présidé par M. Laignel, dans

nous discutons est une négation de l'intercommunalité. L'intercommunalité, ce n'est pas mettre des territoires ensemble ; c'est faire de l'intégration.

Cette mesure a été justifiée par la seule nécessité de respecter un parallélisme des formes avec les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Sur le fond, lorsqu'une communauté de communes n'exerce pas elle-même les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, que ce soit en l'absence de transfert de la part de ses communes membres ou bien dans le cas où ces compétences sont exercées par un syndicat dont cet EPCI fait partie, la minoration de son CIF qui en résultera aura concrètement pour effet de diminuer le montant de sa dotation d'intercommunalité. Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette disposition, adoptée sans aucune concertation ni aucune étude d'impact préalables.

Je précise que la commission des finances de l'Association des maires de France, qui s'est réunie ce matin, estime également que la prise en compte dans le calcul du CIF des communautés de communes du produit des redevances d'eau et d'assainissement à compter de 2020 a été adoptée sans étude d'impact ni concertation.

Cet amendement vise à corriger une erreur. Il s'agit de ne pas décaler l'entrée en vigueur d'une disposition ayant vocation à s'appliquer dès 2019, à savoir la prise en compte des dépenses de transfert dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes à fiscalité additionnelle.

vote. Monsieur le président, ce qui est tout à fait exceptionnel avec la majorité à l'Assemblée nationale, c'est qu'elle ne nous déçoit jamais. On en a toujours pour notre argent ! Quand il n'y en a plus, il y en a encore.

Nous sommes tous ici des élus locaux de longue date. Nous sommes tous des femmes et des hommes qui avons un bilan. Les citoyens de nos départements le connaissent et savent

J'ajoute qu'il faut également veiller à ne pas pénaliser les communautés de communes dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans celui d'un syndicat mixte d'eau et/ou d'assainissement, et qui souhaiteraient préserver ce mode d'organisation territoriale si elles estiment que celui-ci est pertinent a fait les preuves de son efficacité. C'est pourquoi le présent amendement prévoit, dans ce cas de figure, d'exclure les redevances d'eau potable et d'assainissement du calcul du CIF des communautés de communes. Il convient de noter, toutes choses étant égales par ailleurs, qu'un tel dispositif de « neutralisation » existe déjà pour la compétence déchets,

dans celui d'un syndicat mixte d'eau et/ou d'assainissement, et qui souhaiteraient préserver ce mode d'organisation territoriale si elles estiment que celui-ci est pertinent et qu'il a fait les preuves de son efficacité. C'est pourquoi le présent amendement prévoit, dans ce cas de figure, d'exclure les redevances d'eau potable et d'assainissement du calcul du CIF des communautés de communes. Cela a été déjà dit, un tel dispositif de neutralisation existe déjà pour la compétence déchets. J'espère que nous trouverons une solution pour ne pas pénaliser les services d'eau et d'assainissement. J'ai tout de même le sentiment que,, d'aucuns souhaitent tendre vers la suppression des syndicats locaux pour plus d'efficience. L'amélioration du CIF en cas de prise de compétences dans des délais courts pénalisera surtout les communautés de communes qui les prennent et les transfèrent à de grands syndicats, alors que l'objectif est le même. Dans l'absolu, le calcul du CIF

de la ressource en eau, d'autant plus que la gestion des aléas climatiques nous incite à des regroupements, des mutualisations techniques et financières, des interconnexions des réseaux et des ressources qui dépassent les périmètres des EPCI.

Cet amendement vise à tenir compte des attributions de compensation négatives dans le calcul du CIF. La commission est favorable à cet amendement, tel qu'il

communes éligibles à la dotation de solidarité rurale, la DSR, se regroupent et passent le cap des 10 000 habitants, elles deviennent éligibles à la dotation de solidarité urbaine,

et en Anjou. Je propose un effort soutenable, qui ne coûte rien à personne, et qui permettra même de redistribuer aux autres communes une partie de la DSR de ces communes nouvelles.

Il faut quand même reconnaître que ces communes se sont engagées dans une réforme territoriale extrêmement volontariste. Les petites communes qui se sont associées en communes nouvelles restent des communes rurales

en verrons les conséquences, notamment après les prochaines élections municipales. S'il n'y a pas une volonté réelle et partagée par l'ensemble des forces communales

Nous sommes plusieurs sénateurs et sénatrices à porter les amendements de notre collègue Martial Bourquin. Il nous semble indispensable en effet de redéfinir les critères d'attribution des dotations de l'État, notamment la DSU et la DSR. Rassurez-vous, nous ne nierons pas que le Gouvernement travaille sur un projet de réforme fiscale, mais il est des inégalités qui doivent être corrigées au plus vite, notamment à travers ce projet de loi de finances pour Je m'explique : l'entrée de nombreuses petites villes ou communes rurales dans des communautés d'agglomérations ou des communautés de communes plus importantes a eu comme conséquence un effondrement

Elle s'explique notamment par le fait que, pour la DSR par exemple, seuls deux critères sont retenus : le potentiel fiscal par habitant et le revenu moyen par habitant. Le potentiel fiscal par habitant compte pour 70 % dans le calcul de la DSR et plusieurs communes ont vu leur potentiel fiscal augmenter nettement en raison du changement d'échelle intercommunale, alors que leur revenu moyen est resté identique. Ainsi, ces deux amendements visent à rétablir plus d'équité en augmentant le poids du revenu moyen par habitant afin de prendre réellement en compte la précarité existant dans une commune, laquelle nécessite aussi davantage de politiques publiques en direction des personnes fragilisées.

d'une part de CVAE des départements aux régions sur le calcul du potentiel fiscal des départements et des régions. Concrètement, le potentiel fiscal de tous les départements a été réduit de la part de la cotisation Mais comme la CVAE représente une plus forte proportion des ressources dans les départements « riches », leur potentiel fiscal a été plus fortement réduit que celui des départements « pauvres », ce qui a pour effet d'avantager les départements « riches » dans les calculs de péréquation. L'idée de cet amendement est de comptabiliser les attributions de compensation versées par la région comme une ressource fiscale et, à l'inverse, de considérer les attributions de compensation versées par le département à la région comme une ressource fiscale négative. L'objectif est ainsi de corriger l'effet contre-péréquateur du transfert de la CVAE. Cet amendement reprend le dispositif concernant les communes membres d'un groupement à fiscalité propre.

que le potentiel financier pris en considération dans le calcul des différentes composantes des dotations soit fondé sur

les maires et les conseils municipaux qui se sont engagés dans des projets d'investissement ou des politiques publiques à l'égard de leurs administrés. Il y a là une vraie difficulté,

150 millions d'euros. Quand on connaît la totalité des besoins, le reste à charge pour les allocations individuelles de solidarité et l'explosion de la dépense pour les mineurs étrangers isolés, on voit bien que le compte n'y est pas

on parle beaucoup d'autonomie des collectivités. Quand un département accepte de faire un geste pour ses voisins, laissez-le faire

M. Laurent Lafon, pour explication de vote. Mes chers collègues, si vous ne connaissiez pas l'Île-de-France, vous avez cet après-midi un bel aperçu de la situation

que le département qui concentre, avec les Hauts-de-Seine, l'essentiel de la fiscalité régionale ne participe pas à ce système de péréquation.

ami Roger Karoutchi, je suis un éternel optimiste, et j'espère que la métropole du Grand Paris verra le jour. Les Parisiens n'auront plus alors à subir cinq niveaux d'administration territoriale. Normalement, la métropole du Grand Paris aurait dû être mise

pas d'accord entre collectivités pour d'autres choses derrière. Cet amendement, que j'avais déjà présenté l'année dernière, vise à augmenter de 20 millions d'euros le Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, le FSRIF, qui concerne non pas les départements, mais les communes.

Paris verse effectivement 180,3 millions d'euros au FSRIF, pour une population de 2,2 millions d'habitants, soit 80 euros par habitant ; pour les Hauts-de-Seine, où 18 communes sont contributrices, c'est 101 millions d'euros pour 940 000 habitants, soit 107 euros par habitant. Monsieur Féraud, c'est facile de faire porter sur les autres un nouvel effort de solidarité quand on n'y participe pas

à toutes les communes contributrices, comme à toutes les communes bénéficiaires. C'est pour cette raison que je ne voterai pas cet amendement. contre l'idée d'un plafond. Quand on regarde avec un peu de recul l'évolution des recettes fiscales, on voit que les communes les plus riches continuent de s'enrichir et que les communes les plus pauvres continuent de s'appauvrir. L'idée même de plafonner la contribution des communes les plus riches fait que l'écart de richesse

Il vise à réduire des flux entre les collectivités gonflant artificiellement leur budget. Ces flux, où les collectivités ne jouent que le rôle de boîtes aux lettres, ne contribuent pas à la lisibilité de leur situation financière

de l'Île-de-France ! C'est sûr ! S'il était adopté, cet amendement, dont l'objectif est d'améliorer la visibilité des flux financiers entre les EPCI et les communes, se traduirait en réalité par une plus grande complexité, et ne permettrait plus de distinguer ces différents flux, l'attribution de compensations constituant en réalité le solde. Il serait en outre défavorable aux communes en cas de minoration des dotations transférées.

j'estime préférable de ne pas imposer cette dépense supplémentaire à l'État. Dans un élan de sagesse, je retire donc cet amendement.

L'exploitation de ces aires entraîne des coûts de fonctionnement et de réhabilitation importants et disproportionnés par rapport aux moyens des intercommunalités. De plus, l'exploitation de ces aires présente également fréquemment un déficit considérable, qui reste à la charge de la communauté de communes. Je propose donc la création d'une participation de l'État au fonctionnement de ces aires.

à hauteur d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage conventionnée. Il ne me semble pas opportun d'aller au-delà, d'autant que les crédits de cette dotation viendraient, malgré votre demande, en déduction de l'enveloppe globale de la DGF. L'avis est défavorable.

a trait à une question qui se pose dans beaucoup d'intercommunalités depuis que le périmètre des communautés de communes a été élargi. À partir de là, il s'est trouvé des situations où des communes relativement pauvres ont intégré des intercommunalités

avoir un effet très négatif sur le calcul des potentiels fiscaux et financiers d'un certain nombre de communes membres et, partant, sur le montant de leurs dotations, ainsi que sur leur éligibilité aux mécanismes de péréquation des entités dont ces communes sont membres. C'est un phénomène assez général calcul qui a eu lieu a conduit à des évolutions importantes des dotations de certaines communes. On a notamment pu constater que certaines des communes qui avaient été intégrées à des EPCI composés de communes bénéficiant de potentiels fiscaux et de ressources plus importants avaient vu leur propre potentiel fiscal augmenter fortement en 2018, réduisant leurs dotations

de périmètre, d'obliger la collectivité à faire un rapport sur les gagnants et les perdants de l'opération, et que ce rapport fasse l'objet d'une discussion

bien entendu M. le rapporteur spécial et M. le ministre. L'idée de disposer d'un rapport présenté par l'exécutif, qui permette de mettre les choses à plat et d'avoir un bon diagnostic des mouvements ayant eu lieu au sein de l'intercommunalité pour chacune des communes,

dont la DGF peut varier. Si elle varie, c'est tout simplement que les services de l'État appliquent la loi. La pédagogie permet bien évidemment d'expliquer les choses.

dont les périmètres ont été élargis, ont vu artificiellement leur richesse augmenter, alors qu'elles étaient éligibles à la dotation de solidarité rurale, plus exactement à la fraction cible.

que le lissage s'impute sur la fraction de la fameuse DSR

de sortie de la part « cible » de la DSR. Effectivement, il existe aujourd'hui deux mécanismes de garantie de sortie pour les parts « bourg-centre » et « péréquation », mais aucun pour la part « cible ». Les montants de cette dernière ont beaucoup évolué et peuvent représenter des sommes importantes pour les 10 000 communes concernées, par exemple, plus de 250 000 euros pour une commune de Maine-et-Loire. Il apparaît que la modification des périmètres des intercommunalités a des effets directs sur le classement de la part « cible » des communes. En effet, une commune dite « défavorisée », en intégrant un groupement à fiscalité propre dit « riche », voit sa richesse économique communale augmentée fortement par le jeu d'une répartition des montants de produits fiscaux économiques par habitant. Ainsi, le rang d'une commune qui devient artificiellement riche peut chuter au-delà des 10 000 communes les plus défavorisées et cette commune perd immédiatement cette fraction de la DSR. Ce cas de figure est fréquent et rien ne justifie qu'une commune soit exclue de la fraction « cible » de la DSR en raison d'une conséquence non évaluée de la réforme de la loi NOTRe. Il vous est donc proposé de prévoir un mécanisme de garantie de sortie de garantie de sortie pour permettre à ces communes et à l'intercommunalité intégrée de prendre en compte l'ensemble des conséquences de l'évolution des périmètres intercommunaux sur une période de cinq ans.

En 2018, 1 586 communes ont perdu leur éligibilité à la DSR « cible »- ce chiffre s'élevait à 731 en 2017 et à 719 en 2016 -, souvent en raison d'une hausse de leur potentiel financier à la suite d'une modification de la carte intercommunale. La somme des attributions de DSR « cible » perçues par ces communes en 2017 s'élevait à 29,5 millions d'euros, ce qui représentait en moyenne 3,7 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal. En première lecture du présent projet de loi de finances, l'Assemblée nationale a introduit un mécanisme de garantie non renouvelable pour les communes qui perdent leur éligibilité à la DSR « cible » sous la forme d'une attribution égale à la moitié de celle qui avait été perçue l'année précédente. Toutefois, ce mécanisme ne s'appliquera que pour les communes qui perdent leur éligibilité à compter de 2019. Compte tenu du nombre important de communes ayant perdu leur éligibilité à la DSR « cible » en 2018, il est proposé, à titre exceptionnel, de les faire bénéficier en 2019, au titre de 2018, de ce mécanisme de garantie.

rester à la seule métropole du Grand Paris. À l'Assemblée nationale, les députés sont revenus sur ce dispositif et ont instauré un moratoire pour l'année 2019, en changeant dans la loi le « 31 décembre 2018 » en « 31 décembre 2019 ». Mais ils ont souhaité ont souhaité redonner un petit peu de recettes à la métropole du Grand Paris en supprimant l'unique élément de péréquation qui existe aujourd'hui à l'intérieur de la métropole du Grand Paris, à savoir la DSIT, la dotation de solidarité à

en fonction de critères qui prennent en compte, notamment, le potentiel financier et fiscal des communes. Celles dont les besoins sont les plus importants reçoivent le plus cet outil de reversement de la péréquation. Je défends avec d'autant plus de vigueur cet amendement que,

Quel est l'avis du Gouvernement ? Sujet complexe s'il en est ! Tout à l'heure, un sénateur s'est laissé aller à un peu de brutalité dans le langage, en disant que le Président de la République voulait décider tout seul du sort de la métropole du Grand Paris ...

de vote. Monsieur le ministre, vous tentez de donner une vision politique d'une chose qui est beaucoup plus simple et facile à comprendre. Du fait de l'instauration d'un double niveau d'intercommunalité, les communes ont perdu une part de leurs ressources pour faire face à un certain nombre d'investissements. La loi NOTRe a très logiquement

des équipements de développement économique ou des équipements sportifs ou culturels. Or l'Assemblée nationale a revu les choses en supprimant cette DSIT, qui est une aide et un soutien aux territoires,

nous demandons de revenir à une situation plus compréhensible et plus normale dans laquelle les territoires ont l'argent pour financer les compétences qui leur ont été confiées. Cet amendement est très important afin que les territoires ne soient pas pris à la gorge et puissent financer leurs compétences

pour plusieurs raisons. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'organisation actuelle est totalement insatisfaisante. Elle est hybride et inefficace. La vraie solution, c'est une refonte de l'organisation dans un sens ou dans un autre. En tout cas, on ne peut pas rester dans la situation

et de bon sens. En effet, s'il y a des reproches à faire à la métropole, il y en a aussi à faire aux territoires. Un certain nombre d'entre eux ont choisi- c'est leur choix, je ne le remets pas en cause -de transférer peu de compétences et, du coup, d'avoir peu de besoins.

Et les deux territoires qui ont le moins perçu sont deux territoires de la Seine-Saint-Denis : Paris Terres d'Envol et Est Ensemble, à hauteur d'un peu plus de 400 000 euros chacun. On est donc loin d'un outil de péréquation. s'agit d'un outil de compensation, de retour d'une partie de la CVAE vers les territoires sur lesquels elle est générée. Raison de plus ! Je pense, au contraire, qu'on peut faire davantage de péréquation à travers la métropole.

que cette métropole a été créée par une décision du Gouvernement, sous la présidence de François Hollande, par un vote au Parlement, contre l'avis de la plupart des élus d'Île-de-France, lors du débat qui a eu lieu sur le territoire. J'étais, je l'avais dit à la ministre à l'époque, favorable à ce que la région soit la métropole.

qu'il allait faire des annonces. D'ailleurs, à quatre reprises, on a décalé les annonces attendues du Président de la République sur ce qu'il voulait faire de la métropole. Et, gentils comme nous sommes, nous avons attendu, sauf qu'à un moment, on nous a dit :

Attendons de savoir ce que vous voulez faire de la métropole ! Attendons de savoir ce que devient la région ! Qu'est-ce qui change ? Aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien ! Plus aucune commune ne sait ce qu'elle veut

Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur le ministre ! Vous nous avez dit que vous étiez là depuis peu et que vous consultiez. C'est une affaire extrêmement compliquée, je ne dirai pas le contraire. Ce que nous demandons avec cet amendement, c'est le maintien de ce qui a été voté dans les lois NOTRe et MAPTAM, point barre

Le programme du Président de la République comportait la suppression des départements de la petite couronne, une vraie métropole intégrée. Depuis, on ne parle plus de rien et on se trouve avec un texte

Je peux partager l'idée d'une vraie métropole avec lui, mais en tout cas, je ne peux pas accepter l'idée que, sans réforme, on vide les territoires de la seule substance qui est la leur aujourd'hui. Je rappelle que, à l'origine, ils avaient été conçus pour être des entités sans

Ici viennent de parler, Philippe Dallier, ancien vice-président de la métropole du Grand Paris, et moi, qui suis membre de la commission des finances de la métropole du Grand Paris. Je pense que nous savons de quoi nous parlons quand nous venons demander un vrai moratoire ! Pour une fois, faites-le, au moins ici

alors que la loi NOTRe prévoyait son extinction à la fin de cette année, sans aucune compensation, au bénéfice de la métropole du Grand Paris.

Une commune de moins de 10 000 habitants doit pouvoir recevoir, elle aussi, une bonification, juste compensation des pertes de recettes liées à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L'État se doit de reconnaître l'effort de chaque collectivité.

ou, comme ici, environnementale de la commune, il va tout de même falloir procéder au redressement de cette dotation. Ajoutons-y les effets systémiques de la métropolisation, les garanties accordées aux communes nouvelles, et je ne sais quoi encore, et nous voici face à un problème insoluble, qui peut d'ailleurs

parce qu'il faut préserver la nature, ce qui est une très bonne chose ; d'autre part, comme elles ne se développent pas, elles n'auront plus de services, puisqu'on ne sera pas assez nombreux à habiter là. Pour une fois, c'est une bonne solution de montrer que l'écologie peut être vertueuse

Dans certains départements, notamment la Haute-Savoie, toutes les collectivités sont contributrices nettes au FPIC, quelles que soient leurs ressources, en raison de leur caractère frontalier. En effet, elles sont pénalisées par le critère du revenu par habitant, du fait de la présence sur leur territoire

Les corrections nécessaires du potentiel fiscal des communes devraient pour cela découler d'un ordre renouvelé, puisque l'ordre actuel est dépourvu de toute cohérence et de toute logique. Pour le dire autrement, il serait légitime et juste de prendre en compte les effets des différents mécanismes de péréquation horizontale dans le champ du potentiel fiscal. est l'objet de cet amendement. Sans remettre en cause la définition actuelle des potentiels fiscal et financier, nous voulons appliquer pleinement les modalités de calcul du potentiel fiscal pour intégrer tout à la fois les effets des péréquations départementales et régionales, ainsi que les effets liés au FPIC. Les amendements

Or les montants versés correspondent bien à une ressource pour les collectivités concernées. Avec cet amendement, nous en venons à un niveau de complexité que seuls peuvent nous réserver les finances locales et, plus particulièrement, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. L'amendement n° II-676 rectifié étant lié à l'amendement n° II-674 rectifié, je les présenterai en même temps, permettant ainsi à nos débats d'avancer prestement,

sur sa décision de créer deux régimes différents et d'inclure l'outre-mer dans le droit commun. Tous les calculs montrent que nous serons plus avantagés par cette nouvelle péréquation. L'amendement

Monsieur Hervé,

Ce sous-amendement tend à faire en sorte que la commission d'élus puisse donner son avis sur l'ensemble des dossiers présentés. Le sous-amendement n°

alors que seuls des représentants de communes et d'EPCI ruraux siègent au sein de l'actuelle commission DETR. En effet, la nouvelle commission devrait nécessairement être élargie aux autres communes. Les représentants des communes et EPCI urbains interviendraient donc même pour même pour l'attribution de la DETR réservée aux communes rurales. Ces deux dotations sont attribuées par l'État pour financer des projets d'investissement. D'ailleurs, il ne s'agit pas de dotations libres d'emploi, comme, par exemple, la dotation globale de fonctionnement. Nous sommes favorables à une plus grande transparence des subventions attribuées- c'est le sens de l'amendement que je viens de vous présenter -, comme c'était d'ailleurs le cas pour la réserve parlementaire. On ne voit pas pourquoi les préfets ne seraient pas soumis aux mêmes contraintes ou à la même transparence. En revanche, il ne nous semble pas utile de prévoir une nouvelle commission pour assister le préfet qui attribue la DSIL. Les priorités financées par cette dotation sont fixées par la loi. Créer une telle commission risquerait de retarder encore l'attribution des financements.

ne sont pas les mêmes que ceux qui sont éligibles pour la DSIL. Il y aurait donc rupture d'égalité. Il faudrait expliquer à quelques élus, par exemple, dans votre département, d'Évreux, de Louviers ou de Vernon, que les dossiers de DSIL passeraient devant une commission dans laquelle ils ne seraient pas représentés.

commission des lois. Je dois d'abord me réjouir de la qualité du travail que la commission des finances et la commission des lois ont effectué ensemble sur cette matière, qui est évidemment essentielle pour nos collectivités. Je veux aussi remercier M. le ministre d'avoir pris le soin d'expliquer son point de vue de manière très détaillée. Nous voudrions avoir un système plus simple

des communes rurales. Sur le premier point, qui nous paraît très important, que se passe-t-il actuellement ? Nous avons en effet une dotation de soutien à l'investissement local qu'il appartient actuellement aux préfets de région de répartir.

Mais le système est tellement lourd à gérer d'un point de vue administratif que les crédits de la dotation sont en réalité sous-consommés ; au fond, la procédure administrative est beaucoup trop lourde et bureaucratique. À nos yeux,

dans son département de l'attribution de toutes les subventions aux collectivités locales, syndicats intercommunaux et communautés de communes. Instituons donc une commission également compétente pour

vote. Dans le cas où notre assemblée réserverait un sort favorable à cet amendement, un certain nombre d'amendements déposés par notre collègue Didier Marie tomberaient.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi que l'a rappelé en début de séance M. le président de la commission des finances, la conférence des présidents a décidé que la discussion des articles rattachés et des amendements portant sur ces articles